Benbassa, sur l'article. Après de très nombreuses heures passées sur ces travées à étudier la grande majorité des dispositions de ce texte, nous arrivons finalement à l'article qui a causé le plus de controverses dans l'opinion publique et a mis le Gouvernement dans l'embarras, à juste à juste titre. Comment peut-on imaginer que la France, pays des droits de l'homme, puisse renier le plus cher de ses acquis, à savoir la liberté d'expression ? Comment peut-on concevoir que la presse française se retrouve muselée par un État qui ne sait ni regarder ni sanctionner les mauvais comportements de ses propres agents lorsqu'il y a lieu La population sera, par ce texte, soumise à une surveillance généralisée, mais on lui interdira de procéder à des captations d'images susceptibles d'identifier des agents de police et de gendarmerie pour dénoncer des actes de violence policière. Il arrive déjà, en pratique, que les forces de l'ordre s'opposent à ce qu'elles soient filmées ou photographiées en pleine action. Pourtant, une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 23 décembre 2008 précise que cette opposition est contraire au droit. Ce problème, ainsi que l'impunité qui règne parfois dans les rangs des forces de l'ordre et qui sape la relation de confiance qui devrait exister entre les citoyens et celles-ci, aurait dû être abordé dans ce texte, surtout que les infractions contre l'intégrité physique ou psychique des agents sont déjà prévues par le code code pénal. Il aurait en revanche été utile de définir précisément cette notion, ainsi que celle d'impact psychique, qui s'avère aussi floue dans le droit actuel que dans la présente proposition de loi. Comme nous l'avons déjà répété, ce texte est très lacunaire. La parole

la proposition de loi du groupe La République en Marche s'attaquait directement aux journalistes. En effet, c'est la loi de 1881 qui était visée. C'est le fait de diffuser des images pouvant porter atteinte à l'intégrité physique et psychique d'un agent de police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la police municipale qui pouvait être sanctionné d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende. Le tollé fut général et des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour défendre la liberté de la presse et les libertés publiques. La majorité sénatoriale a habilement reculé pour mieux sauter. Vous ne faites plus référence à la loi de 1881, monsieur le rapporteur : vous introduisez dans le code pénal une disposition générale qui pourra- j'insiste sur ce point -concerner les journalistes comme les autres citoyens. le premier alinéa de l'article 226-4-1-1 du code pénal est si limpide qu'elle pourrait passer inaperçue : « La provocation, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la police municipale [ ...] est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » En droit, les mots comptent. Vous ne pouvez pas dire que les journalistes ne peuvent pas être visés par une telle mesure si la justice en décide autrement ! C'est la justice qui décidera si la diffusion d'images relève de la provocation à l'identification ou pas. Pouvez-vous m'assurer que le juge, s'il est saisi de la diffusion d'une image comprenant le numéro d'immatriculation d'un agent, par exemple, ne décidera pas qu'il y a eu provocation à l'identification ? Votre rédaction laisse entière la menace contre la liberté de la presse et renforce fortement les sanctions contre les diffusions d'images. Le parallèle que vous dressez dans votre rapport avec la provocation au suicide, la provocation de mineurs à consommer des stupéfiants ou même la provocation à un assassinat apparaît éculé, outrancier et, surtout,

des poursuites d'ordre général, et pas seulement en matière de terrorisme, contre la diffusion d'images de policiers, gendarmes ou policiers municipaux, entre autres. Nous voterons donc contre cet article 24.

Cet article comporte des mesures sans effet dès lors que des millions de téléspectateurs pourront découvrir le visage des policiers dans leur mission de maintien de l'ordre, trop souvent face à des émeutiers de plus en plus violents, dont les visages n'apparaissent pas à l'écran. Le visage est reconnu comme un élément d'identification. La captation par l'image d'un visage est encadrée par la loi. L'article 24 ne définit pas ce qu'est un élément d'identification, dès lors qu'il exclut le mot « visage ». Il crée une inégalité

Le débat n'oppose pas ceux qui voudraient protéger les policiers et ceux qui ne le voudraient pas. Mes chers collègues, oui, nos forces de l'ordre doivent être protégées quand elles sont attaquées ou menacées, et les familles de leurs membres encore plus. Nous partageons cette préoccupation. Nous n'avons aucune mansuétude envers ceux qui incitent à la haine contre les agents qui font l'honneur de la République. je relève qu'ils sont déjà protégés légalement par la loi de 1881 et par le code pénal. Les policiers disposent d'un arsenal législatif pour lutter contre les menaces, le harcèlement, les atteintes à la vie privée, etc., et c'est heureux. Aucun élément sérieux ne démontre que ces qualifications juridiques seraient insuffisantes. La protection des policiers exige d'abord que ces lois soient appliquées sans faillir. Elle passe aussi par le renforcement du lien de confiance entre la police et la population, et c'est là que le bât blesse. En réalité, ce texte traduit la faiblesse du Gouvernement, qui ne parvient pas à contenir le phénomène alarmant de la multiplication des violences policières.

La moindre professionnalisation ainsi que la réduction brutale des effectifs spécialisés ont conduit à une augmentation massive de la violence. Cette orientation doit être modifiée. 2 500 blessés chez les gilets jaunes, 1 800 chez les policiers, 122 journalistes blessés ou entravés dans l'exercice de leurs fonctions. Ces chiffres ne plaisent à personne- encore moins peut-être aux membres de notre Haute Assemblée ... Ce que nous disons, c'est que la police française se replie sur elle-même, sur ses techniques, sur sa doctrine. Or, dans une démocratie, le niveau de monopole de la violence légitime est établi par l'État. lors que l'État revendique ce monopole, il se doit d'être exemplaire. En démocratie, la liberté, c'est aussi le contrôle citoyen sur celles et ceux qui exercent l'autorité. Je n'invente rien : c'est l'article XV

monsieur le ministre, mes chers collègues, la liberté de la presse est un bien tellement précieux que nous devons y veiller comme à la prunelle de nos yeux.

passé. Nous sommes pour la liberté de la presse totale et intégrale. La loi de 1881, qui n'a jamais été remise en cause, est un bien extrêmement précieux.

mon cher collègue. Il nous reste à supprimer cet article 24 pour défendre la liberté de la presse.

du visage ou de tout élément permettant l'identification d'un fonctionnaire de police, d'un militaire de la gendarmerie ou d'un policier municipal. Je souligne bien entendu le

de l'article 24 fait référence à la CNIL : il prévoit la répression de la constitution de fichiers visant des fonctionnaires et des personnes chargées d'un service public dans un but malveillant. Je soutiendrai bien entendu cet article.

Reprenons cette question : qui, aujourd'hui, chez les fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, a peur d'être filmé ? Je n'ai pas la réponse. Je vous la laisse, monsieur le ministre ... Mardi, vous avez affirmé que les policiers sont les fonctionnaires les plus contrôlés, poursuivis et sanctionnés. C'est bien légitime et heureux ! Leurs responsabilités sont immenses ils ont la possibilité de contrôler, d'interpeller, d'arrêter, d'utiliser la coercition au nom de l'État, dans le respect absolu de la proportionnalité. Il est donc parfaitement légitime que l'usage de ce pouvoir fasse l'objet d'une attention constante, dans un esprit de garantie de nos libertés. C'est pourquoi ces fonctionnaires doivent pouvoir être filmés Donner aux forces de l'ordre les moyens d'empêcher d'être filmées, comme cet article le permettra, jettera la suspicion permanente sur leurs actions. Pourtant, la confiance doit être rétablie. Oui, les images que nous avons pu voir ces derniers mois concernant le maintien de l'ordre ont permis de faire connaître des abus. On ne protégera pas l'institution policière avec des oeillères ! Il faut lutter contre la mise en danger de la vie des agents. Il est temps d'apaiser les esprits et de restaurer la confiance, ce qui passe par une autre doctrine de maintien de l'ordre, l'actuelle étant dans l'impasse. Il est temps d'envisager la désescalade plutôt que la fuite en avant, que cette loi accélère. Mes chers collègues, écoutons nos concitoyens et les journalistes. Laissons-les témoigner. Permettons-leur de rétablir la confiance trop longtemps dégradée. Pour cette raison, nous souhaitons l'abrogation de cet article. La

Le Conseil de l'Europe, qui est, ni plus ni moins, le garant des libertés fondamentales en Europe, nous a exhortés, en décembre dernier, à amender cet article, estimant qu'il portait atteinte à la liberté d'expression.

On ne peut nier que cet article renforcera l'impunité policière et cette propension des forces de l'ordre à s'opposer au fait d'être filmées au cours d'une opération. Même s'il n'interdit pas en soi de filmer, il n'en demeure pas moins qu'il va tout changer sur le terrain et donner un blanc-seing aux forces de l'ordre pour s'opposer toujours plus violemment à la prise d'images. Je vous parlais en préambule de la médaille des colporteurs. Aujourd'hui, cet oeil du peuple, ce sont les caméras. C'est grâce à elles que nous pouvons rendre compte de manquements, alerter, témoigner. Elles participent à la vigilance du peuple. On ne protégera pas les forces de l'ordre en créant des dispositifs de nature à nourrir le sentiment de leur impunité. L'État de droit, monsieur le ministre, ce n'est pas l'État policier. L'État de droit, c'est le droit de surveiller l'État.

La crise de notre République procède aussi d'une distance croissante entre une partie de la population et nos forces de police. Il faut donc renouer la confiance réciproque. Or ce n'est pas en mettant en place des dispositifs qui cachent davantage les réalités et en permettant que les forces de l'ordre, au motif de la provocation à l'identification, puissent s'opposer à des prises d'images que l'on réglera ce problème. ce problème. Tout d'abord, on peut s'étonner que les autorités policières et l'ensemble de l'État ne se soient pas suffisamment mobilisés pour utiliser systématiquement le droit existant, qui devrait pouvoir mieux protéger les policiers quand ils sont réellement menacés. Nous avons tous en tête un certain nombre de drames. Mais, dans le même temps,

Les peines prévues ont été alourdies et ce nouveau délit, introduit dans le code pénal et non dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, s'applique également aux familles des membres des forces Cette rédaction est insatisfaisante. La disposition est définie de manière trop large et ouvre la voie à des interprétations arbitraires, qui pourraient contribuer à entraver le travail des journalistes. Cette disposition porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, car le risque de sanctions, l'obligation de supprimer tout élément d'identification sur les vidéos ou images montrant des policiers et le critère d'intention- vous me le concéderez -sont autant d'éléments de nature à dissuader la collecte d'éléments concernant l'action de la police. En ce sens, cette disposition crée aussi des obstacles au contrôle de l'action des policiers et gendarmes, car les vidéos de policiers ont été essentielles pour dénoncer les pratiques illégales de certains membres des forces de l'ordre et, dans certains cas, permettre l'ouverture d'enquêtes. Soulignons enfin l'avis de la Défenseure des droits,

le maintien de la mention de « but manifeste » de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime continue d'octroyer aux forces de l'ordre une marge de manoeuvre importante et subjective sur leur interprétation de l'intention malveillante. Et si la provocation est pénalement déterminée, la notion d'identification ne constitue pas, en elle-même, un fait punissable. Il paraît donc juridiquement dangereux de faire reposer l'élément matériel de ce nouveau délit sur une non-infraction. En outre, le texte ne précise pas si la provocation

un journaliste, un rédacteur ou une personne sans carte de presse qui filmerait, sur le fondement de la diffusion des images.

conformément à l'article X de la Déclaration des droits de l'homme et aux interprétations successives du Conseil constitutionnel. Je suis sûr

par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat,

qui n'est nullement attentatoire à la démocratie et à la liberté de la presse, c'est parce que j'ai considéré que l'interdiction de la diffusion dans le seul cas d'intentions malveillantes semble d'une application très difficile, car soumise à appréciation subjective

les conditions de service de la douane induisant un danger, de manière à ne pas, si j'ose dire, « arroser trop large

nasse, le « nous ne sommes pas dans le même camp, madame », c'est une doctrine qui vise l'escalade et non pas la désescalade. Sans effets de tribune, sans emphase, nous aurions aimé un texte plus solide,

Cet article était mal né, mais il répondait à une nécessité. Il s'agissait- c'est tout le sens de la nouvelle rédaction

que l'expression de points de vue. Je ne peux m'empêcher, comme nous tous ici, de penser aux hommes et aux femmes qui ont été victimes de l'usage d'images

Monsieur Retailleau, vous m'avez invité à remercier le Sénat, ce que je fais bien volontiers. J'ai beaucoup de respect pour mes illustres prédécesseurs, et singulièrement pour Clemenceau qui passa beaucoup de temps à vouloir exclure le Sénat des institutions, pour finalement y finir ... Il était Vendéen

aux voix l'amendement n° 233. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion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

bientôt cinq mois que les bars, les salles de concert, les théâtres, les restaurants, les cinémas et les clubs sont fermés, sans exception. Les femmes et les hommes qui font vivre ces lieux ont besoin de soutien et de perspectives. Ils doivent nous offrir la lumière au bout du tunnel, celle d'une sortie heureuse et joyeuse de la crise actuelle. Cet article permet à des agents hors service de conserver leur arme dans les établissements recevant du public (ERP). Vous comprendrez aisément que la dernière chose dont nous ayons besoin aujourd'hui c'est de la présence d'hommes armés, sans qu'on le sache, dans les festivals, les bars, les clubs et tous les établissements recevant du public. Ce qui doit être rétabli, c'est un droit à la fête et à la culture.

Monsieur le ministre, au sein même du gouvernement auquel vous appartenez, cette mesure fait polémique. Lors d'une table ronde avec le monde de la scène, le cabinet de la ministre de la culture a confirmé que Mme Bachelot avait personnellement pris position contre cet article, et nous ne pouvons que la comprendre. La mesure prévue par cet article ne va pas dans le bon sens. C'est pourquoi nous souhaitons son abrogation. La parole est à Mme Sylvie Robert,

Son bien-fondé ne repose sur aucun élément tangible ou objectif, mais sur des suppositions, voire sur l'établissement de scénarios alternatifs. S'il est possible d'imaginer qu'un gendarme ou un policier armé hors service puisse aider à la résolution d'une infraction constatée en direct dans un ERP, dans un ERP, on peut tout aussi bien envisager qu'un accident se produise, l'arme pouvant tomber dans la foule, être subtilisée, un mouvement de panique pouvant être déclenché, une falsification de carte de police être opérée. En somme, rien ne prouve qu'un policier armé dans un ERP puisse apporter plus de sécurité. Plus

clés du succès de la relance de ce secteur résidera certainement dans la confiance retrouvée du public. Je ne suis pas certaine que ces dispositions y contribuent vraiment. Enfin, plus fondamentalement, l'article 25 représente un changement de paradigme presque civilisationnel, qui nous rapproche d'autres modèles à mon sens très éloignés de notre culture collective et publique. Nous ne devons pas nous résoudre à banaliser ce sujet, comme nous n'avons pas à confondre le renforcement de la sécurité des Français au quotidien par des moyens effectifs et pertinents et le renforcement de l'illusion sécuritaire, auquel appartient définitivement ce dispositif. Je suis saisi

Depuis les terribles attentats de 2015 et, surtout, depuis l'assassinat de deux policiers à leur domicile dans les Yvelines, les agents des forces de l'ordre peuvent plus facilement conserver leur arme de service en dehors de leurs heures de travail. Dans un sens, cette règle est cohérente avec la présomption de service applicable aux forces de sécurité intérieure et aux militaires. Dans l'esprit des majorités d'hier et d'aujourd'hui qui

contrôlera l'authenticité de la carte professionnelle et, donc, la possibilité ou non d'entrer

je crains que certains d'entre nous ne se soient laissé contaminer par une idéologie de course à l'armement, y compris au sein des établissements recevant du public. La théorie, relayée par les lobbys pro-armes américains, voudrait que, pour lutter contre la violence armée, il faudrait une riposte armée.

aussi réconfortante que dénuée de tout fondement. Non, la présence d'une personne armée n'est pas un facteur protecteur dans ce genre de situation ! Jamais rien ne l'a démontré.

Cette position est partagée par de nombreux professionnels des services d'ordre des lieux recevant du public, y compris les stades, ainsi que par tous les organisateurs des festivals de musique, opposés à une telle autorisation.

Un tel dispositif est inquiétant dans la mesure où, en plus de prévoir une autorisation idéologiquement contestable, il n'est pas assorti des garanties nécessaires et suffisantes. Lorsqu'ils ne sont plus en service, les agents de police et les militaires de la gendarmerie doivent pouvoir rejoindre la société civile et s'y mêler dans l'indifférence, d'autant que le bénéfice de leur armement est moins évident à identifier que l'inquiétude et les risques qu'il susciterait. Comment imaginer qu'un agent hors service puisse être armé dans un débit de boissons ?

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

l'a dit. En tant que conseiller municipal et ancien maire de secteur à Marseille, je mesure la responsabilité qu'induit cette disposition. Cependant, le risque terroriste est présent partout, et nous sommes au niveau de vigilance « urgence attentat ». C'est pourquoi je propose l'élargissement du port d'arme hors service aux policiers municipaux habilités à porter une arme. Mercredi 10 mars dernier ont été arrêtés deux islamistes de 17 et 18 ans, dont un à Marseille, alors qu'ils préparaient des opérations sanglantes sur notre sol. Le terrorisme islamiste est alimenté par une politique d'immigration massive et incontrôlée. Il est en partie financé par les réseaux de trafic de drogue. Il recrute dans toutes les couches sociales des hommes, mais aussi des femmes, comme on a pu le constater, de plus en plus jeunes. Cette réalité prouve que la menace va perdurer encore longtemps et se diversifier géographiquement, tant le terreau de notre République, avachie ... Avachie ? ... et affaiblie, est fertile. Nul ne peut imaginer que l'on se prive demain d'agents dûment habilités à être armés et capables de répondre, au même titre que les policiers et gendarmes nationaux, à une menace terroriste réelle qui pourrait se présenter à eux en dehors de leurs heures de service. Ce que les policiers municipaux ont fait à Nice durant leur service, à l'occasion de l'attaque meurtrière d'un pseudo-réfugié, mais vrai clandestin, tunisien, tous les policiers municipaux de France doivent pouvoir le faire si la situation l'impose, Cette disposition que je vous propose est un signal fort envoyé tant aux criminels qu'à nos compatriotes, qui sont évidemment demandeurs de protection. Ils sauront que, désormais, force restera à la loi partout où un représentant des forces de l'ordre se trouvera, en service ou pas. permettra de réaffirmer l'autorité des policiers municipaux et contribuera à endiguer les phénomènes de violence, de barbarie et d'ensauvagement.

Elle prévoyait déjà l'autorisation du port d'arme aux agents de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie nationale au sein d'établissements ouverts au public. Cet amendement ajoute donc un élément de cette proposition de loi, qui prévoyait de devancer les possibles falsifications des cartes professionnelles, en proposant un enregistrement de l'identité des fonctionnaires sur un portail national, dont les modalités d'application seraient fixées par un décret en Conseil d'État. Cette mesure permettrait, en plus d'éviter des usurpations d'identité, d'insister sur la responsabilité de nos forces de l'ordre, qui auront cette démarche supplémentaire à réaliser pour pouvoir délibérément accéder à l'ensemble des ERP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

? Dans un objectif de pacification de la société, il ne nous semble pas pertinent de permettre aux policiers et aux gendarmes de faire usage de leur arme sans être revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité. Il est nécessaire que les policiers et les gendarmes puissent être identifiables ès qualités afin de ne pas provoquer de mouvements de panique. Dans les faits, c'est assez simple pour eux, car il suffit, lorsqu'ils portent une arme, qu'ils disposent également dans leur poche d'un brassard « gendarmerie » ou « police », qu'il leur est facile d'arborer. L'avis est donc défavorable.

normales de service. Cela présenterait un avantage à la fois numérique et stratégique. Premièrement, un tel dispositif permettrait de multiplier à coût zéro le nombre d'hommes entraînés et armés capables d'intervenir immédiatement en cas d'attaque terroriste. Cela a déjà été dit, y compris par vous, monsieur le ministre, en rappelant l'affaire du Bataclan, où, effectivement, un commissaire de police a permis de sauver de nombreuses vies en intervenant. Secondement, la présence aléatoire de militaires dans le cadre de leurs déplacements personnels, en tout lieu du territoire, permettrait de répondre à l'imprévisibilité des attaques terroristes et d'inverser l'effet de surprise à notre avantage. Dans la mesure où policiers et gendarmes sont légalement autorisés à porter leurs armes de dotation et à en faire usage en dehors de leur service, aucun principe ne s'oppose à ce que ce bénéfice soit étendu aux militaires non gendarmes sur le territoire national.

Rappelons que la légitimité du port d'arme en dehors du service par les gendarmes est tirée de l'article L. 4121-5 du code de la défense, aux termes duquel « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

eux-mêmes. Avec le présent amendement, nous proposons que les militaires soient autorisés à ouvrir le feu exactement dans les mêmes cas de figure que les policiers et gendarmes, en dehors de leur service, et selon les mêmes modalités d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité que celles auxquelles ces derniers sont soumis en application des jurisprudences nationale et européenne.

désencerclement, qui ne défendent personne, pas même l'image des forces de l'ordre. L'usage de ces armes est avant tout un mésusage. Les agents, nous le savons, ne sont pas suffisamment et correctement formés à leur utilisation ou, quand ils le sont, ils ne sont pas formés aux missions de maintien de l'ordre. Si nous devions raisonner cyniquement, nous pourrions remarquer que l'utilisation récurrente et outrancière de ces armes n'a qu'un effet très limité, voire contre-productif sur le déroulement des manifestations. En revanche, les revanche, les conséquences physiques et humaines sont gravissimes. Je me permets de rappeler ici la demande de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe de

représente-t-il un tel danger pour le pouvoir en place qu'il faille le réprimer de la sorte ? Les stratégies du Gouvernement portent-elles à ce point leurs fruits que nous devons maintenant discuter de mesures visant à protéger les forces de l'ordre ? Mes chers collègues, puisque cette proposition de loi nous enjoint de penser un continuum de sécurité, pensons ensemble à nos doctrines de maintien de l'ordre et engageons une réflexion sur les stratégies possibles de désescalade. Plutôt que de surarmer consciencieusement tous les agents, de laisser la porte ouverte à une technologie sans limites, nous vous invitons à penser un continuum d'alternatives pacifiques pour nos quartiers, nos villes et pour toutes celles et tous ceux qui y vivent. Tel est le sens de notre amendement.

pour remédier à la culture de l'impunité, qui porte atteinte à l'image des forces de l'ordre et contribue à saper le lien de confiance nécessaire entre celles-ci et la population.

dangerosité : mains arrachées, citoyens éborgnés, manifestants tués. Le Défenseur des droits, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et même Jean-Michel Fauvergue, auteur de la présente proposition de loi, demandent clairement leur interdiction dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre.

réglementée que par des circulaires et des directives du ministère de l'intérieur. Par conséquent, il échappe au législateur. Nous n'avons donc pas pu déposer d'amendement pour l'interdire. Je sais que cela vous embête, monsieur le ministre, mais le rôle des parlementaires est aussi de contrôler l'action du Gouvernement. Aussi, je vous demande solennellement d'interdire une bonne fois pour toutes cette pratique. Vous avez annoncé en juin vouloir en supprimer l'apprentissage dans les écoles de formation. Il me semble que ce n'est pas suffisant. Amadou Koumé, Cédric Chouviat, George Floyd : la liste des victimes est longue. En France, aux États-Unis et partout où il est autorisé, le placage ventral tue ! Depuis 2007, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle la France à l'ordre. Que de temps perdu Pour rétablir la confiance entre la population et sa police, mettons fin à ces pratiques mortelles. C'est d'autant plus important qu'avec ce texte nous transférons des compétences d'interpellation aux polices municipales, et ce sans formation suffisante. Ne perdons pas de vue la mission première du maintien de l'ordre : assurer un cadre apaisé et protecteur pour l'expression légitime de contestations et garantir nos droits à manifester. Je

évidemment une protection générale des policiers et des gendarmes, qui sont plus que tout autre en lien avec l'autorité judiciaire.

d'optimiser l'appui et le support essentiels que représentent les réservistes, afin de renforcer les effectifs de nos forces actives. Il vise à valoriser les compétences des réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et de la gendarmerie nationale, afin de suppléer le personnel actif dans certaines tâches et de faciliter sa mobilisation sur le terrain. La réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et la réserve civile de la police nationale rassemblent des retraités de ces deux corps. Ce vivier démultiplie les forces sur le terrain et renforce leurs capacités, grâce à l'intervention de ce personnel réserviste déjà formé et pouvant être armé. Actuellement, les retraités réservistes qui avaient la qualité d'officier de police judiciaire n'obtiennent que l'habilitation d'agent de police judiciaire, ce qui a pour conséquence de limiter l'utilisation et l'optimisation de leurs compétences, pourtant si utiles sur le terrain. Le présent amendement tend à permettre à ces retraités réservistes anciens officiers de police judiciaire de conserver leur qualité d'officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de leur départ à la retraite. Cette mesure vise donc à augmenter le nombre d'officiers ainsi qu'à augmenter l'efficacité de la réserve civile de la police nationale et des réserves opérationnelles de la gendarmerie nationale. La parole est à M. Henri Leroy, pour

des corps actifs de la police nationale, et non aux personnes justifiant d'avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité. En second lieu, il vise à instaurer une actualisation obligatoire des connaissances pour les anciens OPJ,

C'est pour contribuer à combler ce vide et dans le but de protéger nos forces de l'ordre que je propose, par cet amendement, d'instaurer à l'article 122-6 du code pénal une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre qui font usage de leur arme dans l'exercice de leurs fonctions. Mieux vaut un bon exemple que de longs discours. Ainsi, le dimanche 28 avril 2019, à Marseille, un homme déjà connu des services de police fuyait un contrôle de la police municipale. Après avoir percuté plusieurs véhicules, l'individu chargeait en marche arrière les policiers. Ces derniers, en danger immédiat, ont fait feu pour protéger leur vie et neutraliser le conducteur, geste véritablement héroïque, d'autant que les policiers ont même prodigué les premiers soins au délinquant, lui sauvant la vie ! Dans la plupart des pays du monde, ces hommes seraient décorés et remerciés, mais pas en France ! Dans notre pays, ils sont mis en examen et gardés à vue pendant quarante-huit heures, alors même qu'ils ne présentaient aucun danger de se soustraire à leurs obligations judiciaires et que leurs états de service étaient irréprochables. La situation est ubuesque et scandaleuse, à une époque où nos policiers sont devenus des cibles aussi bien pour les terroristes islamistes que pour les milices d'extrême gauche. Il convient de noter qu'après un non-lieu rendu par le juge d'instruction le parquet a scandaleusement fait appel et demandé le renvoi des deux fonctionnaires devant le tribunal. La protection juridique des forces de l'ordre doit être renforcée ! De plus, alors qu'une sinistre mode venue des États-Unis et largement reprise par certains mouvements et partis de gauche et d'extrême gauche voudrait imposer dans le débat public les termes de « violences policières » et de « racisme systémique

est ainsi libellé : La parole est à M. Pierre Laurent. La politique de sécurité globale envisagée par le présent texte engage dans le continuum de sécurité de nombreux agents supplémentaires : police nationale et gendarmerie nationale, mais aussi polices municipales et entreprises de sécurité privée. Or, pour encadrer le nouveau continuum de sécurité qui nous est proposé, aucun contrôle supplémentaire de l'action des forces de sécurité n'est prévu dans ce texte, si ce n'est une réflexion future évoquée dans le cadre d'une demande d'habilitation à légiférer à légiférer par voie d'ordonnance au sujet des organismes censés veiller au bon déroulement des missions des agents de sécurité privée. Nous estimons pour notre part qu'il est indispensable que des autorités indépendantes exercent, dans le cadre de leurs interventions en matière de sécurité publique,

Il s'agirait de proposer un vrai pouvoir de contrôle et de mise en oeuvre des sanctions si les faits l'exigeaient. Nous ne pouvons aller totalement au bout de notre proposition, article 40 de la Constitution oblige. Nous demandons donc que, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'opportunité de créer pour chaque corps de métier disposant de prérogatives de sécurité publique une autorité indépendante. À chaque occasion, un droit de saisine serait ouvert pour nos concitoyennes et nos concitoyens ; la transparence de ces procédures serait assurée. Quel

: La parole est à M. Philippe Tabarot. Cet amendement a pour objet la sécurisation des transports en commun. Le recours à des agents de sécurité fournis par des sociétés privées de sécurité est possible et fréquent dans le secteur des transports publics, à des fins de gardiennage, de surveillance des emprises et des véhicules de transport, ainsi que de sécurisation des personnes qui les fréquentent, y compris au service des sociétés publiques de transport disposant de services de sécurité internes, comme la SNCF ou la RATP. Les missions de ces sociétés s'inscrivent dans une chaîne de sécurité qui va de la prestation d'agent de médiation intervenant dans les emprises, les haltes et les véhicules de transport apaiser des litiges et soulager le personnel d'exploitation, comme chauffeurs ou contrôleurs, à des prestations de service dissuasives ou actives en appui d'opérations de contrôle ou de sécurisation des usagers. Le recours à des services d'agents de sécurité dans les transports publics, au-delà des forces de l'ordre, ne fait pas l'objet de dispositions distinctes du droit commun. Cet amendement vise donc à clarifier les possibilités laissées aux opérateurs de transport et à autoriser les agents de sécurité privée à disposer du pouvoir d'enjoindre de descendre d'un véhicule de transport et de sortir d'une emprise telle qu'une gare routière, ou encore d'interdire l'accès à un véhicule de transport aux personnes fraudant dans les transports, compromettant la sécurité des passagers, nuisant à la régularité des circulations, ou encore troublant l'ordre public. Outre le renforcement de solutions technologiques innovantes, la présence humaine sur le terrain, dans les véhicules et dans les gares, reste un moyen efficace pour atteindre les objectifs de tranquillité publique. Pour donner aux opérateurs de transport, sur tous les réseaux qu'ils exploitent, les moyens d'assumer pleinement leurs obligations légales et d'assurer la sécurité de leurs voyageurs et de leur personnel, il est impératif de leur laisser le choix de disposer d'un service interne de sûreté ou de faire appel à une entreprise de sécurité privée, en leur permettant d'agir. la commission ? Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux agents de sécurité privée d'enjoindre aux personnes se trouvant en infraction aux règles de transport de quitter les véhicules de transport ainsi que les espaces affectés au transport public. Je sais que c'est une demande extrêmement forte des opérateurs de transport, mais je suis au regret de vous dire, mon cher collègue, que je me dois d'y être défavorable, et ce pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel encadre strictement l'exercice de prérogatives d'ordre public, telles que l'éviction, en particulier lorsqu'elles sont dévolues à des agents de sécurité privée. Ainsi, le pouvoir d'éviction est aujourd'hui réservé aux services de sécurité internes des agences de transport public, ainsi que, le cas échéant, aux officiers de police judiciaire, qui sont spécialement formés et disposent d'une expérience à même de justifier l'exercice de prérogatives spécifiques. Il ne me paraît pas opportun de confier à des agents privés un tel pouvoir d'injonction, qui plus est dépourvu de toutes garanties. Au surplus, cette absence de garanties m'interroge et risque de poser une difficulté d'ordre constitutionnel.

l'ensemble des outils qui leur permettront d'assurer leurs missions face à l'accroissement de la violence et de la criminalité qui touche chaque secteur de la société. À ce titre, et afin que ces forces puissent collaborer encore plus efficacement avec les forces régaliennes dans le cadre du continuum de sécurité, je sollicite l'adoption d'un certain nombre de mesures nécessaires pour une coproduction de sécurité de haut niveau, qui viennent compléter la loi Savary-Leroux. Les agents des services internes de sécurité sont des acteurs incontournables, qui doivent pouvoir continuer, chaque jour, à mettre leurs exigences de qualité de service et de professionnalisme au service des voyageurs et des transporteurs. Cet amendement vise à donner accès aux fichiers des documents d'identité aux agents de sûreté assermentés et agréés des transporteurs, dans l'objectif de soulager les forces de police, qui sont systématiquement sollicitées pour venir contrôler l'identité de voyageurs en infraction. Un accès aux fichiers des documents d'identité pourrait être autorisé pour des agents du service interne de sûreté spécialement habilités et agréés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, afin de procéder aux vérifications. Cela permettrait également d'éviter énormément de retards dans nos transports en commun. commun. Actuellement, un voyageur contrôlé pour absence de titre de transport qui refuse de décliner son identité impose aux agents de la RATP ou de la SNCF de faire appel à un équipage de police, qui doit se déplacer pour procéder à la vérification de l'identité. Il convient donc d'admettre que cette démarche engendre pour la police une réelle surcharge d'activité. La question se pose alors de permettre aux agents de sûreté, ainsi qu'à la police municipale dans le cadre de ses missions dans les transports en commun, d'accéder aux fichiers relatifs aux documents d'identité mis en place, qui permettrait aux forces régaliennes de se concentrer sur d'autres missions. Il conviendrait donc, lors d'une verbalisation, de distinguer le cas où le contrevenant refuse purement et simplement de justifier de son identité de celui où il est simplement dans l'impossibilité de le faire. Une telle opération éviterait de mobiliser la police sur une tâche pouvant être effectuée par d'autres agents et ferait par ailleurs gagner du temps aux agents verbalisateurs sur le terrain.

de faciliter la lutte contre la fraude, qui occupe une place centrale dans la mission de prévention des agents du service interne de sécurité de la RATP et de la SNCF, et de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Faciliter les opérations de verbalisation des contrevenants sur le terrain me paraît essentiel.

je me dois de vous appeler à la prudence sur ce point. En effet, la jurisprudence de la commission des lois est très claire : tout accès aux fichiers doit être justifié au regard des prérogatives dévolues aux agents et des finalités de traitement. Aucun accès direct aux fichiers d'identité pour les agents des services internes de sécurité ne peut être envisagé, car il ne saurait

M. Philippe Tabarot. Au regard de la nature de la criminalité- agressions avec armes -et de la menace terroriste, il conviendrait de faciliter et de rendre plus efficiente la mise en oeuvre des palpations préventives des réseaux (GPSR) de la RATP, en supprimant les exigences d'habilitation et d'agrément, ainsi qu'en permettant un recours à ces palpations, avec le consentement exprès des personnes, en dehors de tout arrêté, dès lors qu'il est constaté sur la base d'éléments objectifs qu'une personne est susceptible de détenir un objet présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. Ainsi, les exigences d'agrément et d'habilitation paraissent superflues au regard du niveau de formation des agents du GPSR et des nombreux contrôles dont ils font l'objet. pour les vols à la tire, les agents du GPSR sont soumis à une liste exhaustive de stations où les palpations peuvent être pratiquées. Si les délinquants se déplacent dans une station voisine non prévue dans l'arrêté, cette prérogative ne pourra pas être mise en oeuvre. Dans un souci d'efficacité dans la mise en place de cette mesure, qui répond plus que d'autres à un sujet de sécurité publique, il convient, à travers cet amendement, de faciliter la mise en oeuvre de ces palpations.

Il conviendrait ainsi de faire évoluer les textes et d'intégrer les agents de sûreté de la RATP et de la SNCF aux catégories de personnels pouvant accéder, dans le cadre spécifique de leur mission, aux informations figurant au sein des passeports, des cartes nationales d'identité des ressortissants français et des cartes de séjour, en réservant cependant cette faculté à ceux qui sont présents dans le PC Sûreté, par exemple.

de la sécurité des transports et les contrôleurs dans leur quotidien difficile. Le secteur des transports est frappé de plein fouet par la pandémie, et la montée de l'insécurité n'incitera certainement pas nos compatriotes à reprendre les transports en commun

et du groupe unifié pour davantage de sécurité juridique, notamment dans le cadre des évolutions liées au réseau du Grand Paris et à la mise en concurrence progressive du réseau historique de la RATP. Quel est l'avis de la commission ? À la

Certes, il nous est dit que l'expérimentation serait limitée au seul transport ferroviaire et précaution est prise de faire expressément référence à la CNIL. Pour

soutenons le déploiement, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, d'un système de vidéoprotection embarqué sur les matériels roulants, dont le but est d'assurer la prévention et l'analyse des accidents de transport. Toutefois, la CNIL s'est montrée réservée sur le contenu de cet article, relevant que, « à défaut « à défaut de précision, la Commission s'interroge sur les conditions ayant conduit à considérer que l'expérimentation menée devait permettre un enregistrement permanent, quand bien même l'exploitation ultérieure des images collectées

jours correspondent à la durée standard de tous les autres régimes de captation d'images. Cet article autorise les opérateurs de transport à équiper leurs véhicules de caméras embarquées afin de lutter contre les accidents, sous la forme d'une expérimentation,

Nous tenons à souligner l'effort qui a été fait par la commission pour limiter le risque d'inconstitutionnalité de cet article. Nous continuons cependant de

lors, pour préserver le droit à la vie privée des usagers des services de transport, tout en répondant aux demandes des exploitants, la commission a exigé de conserver un caractère circonstancié à la transmission des images. Toutefois, elle a accepté d'assouplir légèrement cette condition pour faciliter l'intervention des forces de l'ordre. Ainsi, la transmission doit être possible dès que les circonstances font redouter la commission d'une atteinte aux biens ou aux personnes. En revanche, elle doit continuer à être limitée au temps nécessaire aux services de police pour leur intervention, ou pour la levée de doutes.

vous le souhaitez. Quel est l'avis de la commission ? L'amendement du Gouvernement tend à modifier le dispositif de fiabilisation des données de recouvrement des PV de fraude dans les transports. Il vise à inscrire dans la loi que l'interface entre les agents

Les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF peuvent, à titre expérimental, procéder à l'enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Il est Il est proposé d'étendre cette expérimentation aux agents de sécurité privée qui agissent pour le compte de ces opérateurs de transport.

Autoriser les caméras mobiles de façon générale pour l'ensemble des agents de sécurité privée opérant dans le secteur des transports poserait des problèmes d'ordre juridique. Seuls les agents de la SUGE et du GPSR

La commission a souhaité renforcer cette possibilité pour les agents assermentés par une expérimentation strictement encadrée, qui doit être menée à son terme avant que ne soit étudiée l'opportunité de l'étendre aux agents privés des entreprises de transport. La commission

prévoit qu'un décret en Conseil d'État définit les modalités d'utilisation des données collectées dans le cadre de l'usage des caméras-piétons par les agents assermentés des entreprises de transport. Au regard de l'objet de ce décret, il paraît nécessaire de préciser que celui-ci sera pris après avis de la CNIL.

proposé que les agents de police municipale puissent constater les contraventions découlant de ces contrôles aux fins de garantie. Il est précisé que les agents rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire, de la police nationale ou de gendarmerie territorialement compétent.

326 rectifié vise à rétablir la simplification des modalités de contrôle de l'alcoolémie en l'absence d'infraction. Comme je l'ai souligné en commission, il ne me paraît pas souhaitable de permettre la réalisation d'un éthylomètre sans éthylotest préalable pour tout contrôle routier inopiné.

n° 206 rectifié . Monsieur le rapporteur, que la police municipale puisse procéder aux vérifications d'alcoolémie, s'affranchissant ainsi du préalable de contrôle, est tout de même une amélioration considérable dans l'action des polices municipales, au regard des techniques nouvelles qui sont à disposition et qui doivent être inscrites dans l'ordre législatif.

La disposition prévue à cet amendement fait suite à un entretien que j'ai eu ces dernières semaines avec les brigades vertes du Haut-Rhin. Comme vous le savez, les gardes champêtres jouent un rôle très important en zone rurale. Je tiens à rappeler que c'est lors de la loi de décentralisation de 1988, un amendement du sénateur du Haut-Rhin Henry Goetschy, qu'un regroupement de collectivités réunies en un syndicat mixte a été autorisé dans le but qu'elles aient en commun des gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes adhérentes. C'est alors que les gardes champêtres du département du Haut-Rhin se sont constitués en un véritable corps, aujourd'hui dénommé « brigades vertes », véritable spécificité alsacienne.

Les gardes champêtres accomplissent un travail essentiel de défense des intérêts ruraux. C'est une véritable police de proximité complémentaire de la gendarmerie et de la police. Je souligne aussi le rôle social et relationnel essentiel des gardes champêtres, qui sont de véritables médiateurs ruraux dans les différents litiges. Ils réalisent plusieurs milliers d'interventions chaque année. L'activité relative au code de la route est une grande partie de leur activité. Or ils ne peuvent effectuer les contrôles relatifs aux produits stupéfiants, alors qu'ils peuvent le faire concernant l'alcoolémie. Les gardes champêtres demandent donc une évolution de leurs prérogatives. L'usage de produits stupéfiants au volant est aussi un fléau en zone rurale, notamment chez les jeunes. De plus, le cocktail drogue-alcool multiplie par vingt-neuf le risque d'accident mortel. La drogue circule aussi dans nos communes rurales, ce n'est pas propre aux grandes villes. Au-delà d'un aspect juridique, cet amendement a aussi une portée symbolique. Il s'agit de reconnaître l'action essentielle de nos gardes champêtres dans nos communes rurales pour la sécurité routière et le respect du code de la route.

l'amendement n° 244. Cet article élargit les catégories d'agents publics ou privés habilités à constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du code de la route. du code de la route. Il précise ainsi les infractions qui pourraient désormais être constatées par les gardes particuliers assermentés, notamment des règles concernant la circulation et le stationnement des véhicules. il se trouve qu'ils vont assumer ainsi une mission générale de sécurité publique, au-delà des attributions spécifiques particulières prévues pour ces catégories. Pour cette raison, nous demandons la suppression de cet article, qui concernerait tout de même près de 50 000 gardes particuliers assermentés.

cet article nous semble en partie superfétatoire, incomplet en pratique et ne nous paraît pas répondre à l'exigence de proportionnalité. La limitation du champ territorial d'intervention des gardes particuliers est déjà assurée par l'agrément préfectoral, qui spécifie les limites des droits dont dispose le commettant, à savoir les terrains de l'employeur. En outre, le texte ne prévoit pas le cas de pluralité de commettants, le garde particulier pouvant être commissionné pour plusieurs territoires différents. Enfin, le garde particulier n'est pas un agent de la force publique. Il est d'abord placé sous l'autorité de son employeur- président d'association, de société ou particulier. Il n'a pas pour mission d'assurer la sécurité publique et n'est pas formé pour assurer ce type de mission. Nous préférons en rester au droit en vigueur, aux termes duquel les gardes particuliers disposent d'une compétence judiciaire pour la mise en oeuvre de certaines polices spécialisées dont ils assurent le respect sur le territoire des propriétés qu'ils ont la charge de garder.

libellé : La parole est à Mme Nathalie Delattre. Les gardes particuliers assermentés effectuent une mission essentielle de protection du patrimoine naturel. Ils sont actuellement plus de 12 000 en France. De plus en plus de collectivités territoriales, conseils départementaux, conseils régionaux ou encore établissements publics de coopération intercommunale, recrutent ou commissionnent ces gardes particuliers. Malheureusement, ces derniers ne disposent pas des moyens nécessaires pour répondre aux missions qui leur sont confiées. Pour exemple, le délai imposé de transmission des procès-verbaux est trop contraignant et nuit aujourd'hui à la qualité des procédures engagées. En effet, depuis une ordonnance du 12 juillet 2012, le délai de transmission au procureur a été malencontreusement raccourci à trois jours à compter de la constatation des faits. Or les gardes particuliers sont souvent amenés à procéder à un recueil d'informations de localisation précis concernant le lieu de l'infraction auprès de l'administration compétente, ce qui prend du temps. Il s'agit donc de prévoir que ce délai s'applique à partir de la clôture, et non plus du jour de la constatation de l'infraction. Quel

afin que celui-ci soit la date de clôture du procès-verbal. Ce changement ne nous paraît pas opportun. En effet, seule la mise en oeuvre de pouvoirs d'enquête, susceptibles de durer dans le temps, justifie que le point de départ du délai de transmission des procès-verbaux soit fixé au jour de la clôture du procès-verbal. Tel n'est pas le cas des gardes particuliers assermentés, qui ne mettent pas en oeuvre des pouvoirs d'investigation. Pour ces raisons, la commission demande le retrait

en veillant au respect des espaces qui sont sous leur protection. Ils contribuent également à veiller à la tranquillité de la faune sauvage, qui, nous le savons, est de plus en plus menacée. Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser les circulations et les stationnements interdits dans les espaces boisés. Cette disposition demande à être élargie aux espaces non boisés, où ils relèvent également des atteintes, mais ne sont toujours pas habilités à les sanctionner. Il paraît donc nécessaire de corriger cet écueil, tant pour les gardes particuliers assermentés exerçant dans les collectivités territoriales que pour ceux qui sont employés par des propriétaires privés. Quel

non boisés comme dans les espaces boisés. L'amendement vise à prévoir un strict encadrement des prérogatives avec champ territorial expressément prévu et champ contraventionnel limité à la verbalisation des infractions en matière de circulation, arrêt et stationnement pouvant être interdits dans ces espaces. Par conséquent, la

deux ajouts importants de la commission, qui visent à mieux encadrer les modalités d'enregistrement des données collectées par les opérateurs économiques au cours de l'achat d'articles pyrotechniques, articles en vente libre en application des textes européens. Pour améliorer la traçabilité des achats, il est nécessaire de prévoir de tels dispositifs. La commission des lois a souhaité permettre aux seuls agents publics

est de prévenir les accidents causés par les tirs d'artifice et de divertissement manipulés par des particuliers, mais également d'éviter un détournement de leur usage à l'encontre des forces de sécurité intérieure. Des cas de mutilations pour les forces de l'ordre pour les particuliers- récemment, un jeune homme est décédé en Alsace -exigent de mettre en oeuvre une réglementation plus stricte concernant les tirs d'artifice et de divertissement. Force est de constater que les réglementations successives n'ont pas permis d'éviter ces conséquences dramatiques, notamment pour un public jeune qui les utilise lors d'événements festifs et en détourne parfois l'usage initial. Cet amendement vise par conséquent à compléter compléter le dispositif existant en aggravant les peines prévues en cas d'achat par des particuliers d'articles pyrotechniques en méconnaissance des exigences prévues par la réglementation. Il s'agit non pas d'interdire cette pratique, mais de l'inscrire dans un cadre plus strict, afin de protéger le public, d'une part, et les forces de sécurité intérieure, d'autre part. Ainsi, il est prévu de fixer à six mois d'emprisonnement et à 7 500 euros d'amende 7 500 euros d'amende la vente de ces engins en violation de leur condition d'utilisation, peine doublée si cela est fait par internet, et de fixer à un an d'emprisonnement et à 9 000 euros d'amende la violation des obligations afférentes à ces engins, peine doublée si l'acquisition est réalisée par internet.

les feux d'artifice faisaient rêver les enfants et rassemblaient les générations lors de la fête nationale du 14 juillet ou d'événements festifs. C'était l'époque où l'on tirait à la verticale. Ça, c'était avant

aujourd'hui, une simple intervention policière peut entraîner un déversement de projectiles pyrotechniques d'une violence inouïe. Il semble que l'idéologie du vivre ensemble parte en fumée avec cette nouvelle mode des mortiers d'artifice. dernier, nous découvrions la commune de Champigny-sur-Marne, devenue célèbre pour avoir vu son commissariat se faire attaquer pendant plus d'une heure aux mortiers d'artifice, sans pouvoir intervenir. Au mois de décembre, les images de Chanteloup-les-Vignes ont choqué la France des policiers ont été pris pour cible, les vitres de leur voiture ont volé en éclats, et trois fonctionnaires de police ont été sévèrement brûlés, tout cela pour avoir commis le crime de porter l'uniforme de la police française. Ces violences ont également éclaté aux Mureaux, à Plaisir, à Fontenay-le-Fleury et se propagent maintenant dans toute la France. La semaine dernière, c'était dans le Maine-et-Loire, c'était en Gironde, c'était en Seine-Maritime. Au mois de février, c'est à Poissy qu'une vidéo montrait des jeunes canarder les policiers aux cris de « Tuez-les ! » L'objet de cet amendement est de donner des armes à la justice, d'endiguer un phénomène d'ensauvagement notable, en réprimant plus fortement la récidive. Hier, les voyous attaquaient nos policiers en leur jetant des pierres ; aujourd'hui, ce sont des feux d'artifice. Quelle sera la prochaine étape ? À Marseille, on a déjà la kalachnikov en plein jour dans certaines cités Il faut d'urgence que la peur change de camp, avant que la situation ne nous échappe définitivement et que nos compatriotes, de guerre lasse, ne décident d'assurer eux-mêmes leur sécurité. À la violence des racailles, répondons par l'intransigeance pénale

sont des instances précieuses de dialogue et d'échange entre les acteurs locaux de la sécurité. Ils sont appréciés par les élus locaux et contribuent à l'ancrage territorial de la sécurité et à la fluidité de l'information. nous avons proposé la possibilité d'étendre l'obligation de création des CLSPD aux communes comptant entre 5 000 et 10 000 habitants.

pense que la désignation obligatoire d'un coordonnateur des travaux du CLSPD dans les communes de plus de 10 000 habitants, introduite par l'Assemblée nationale, nationale, n'est pas opportune. C'est donc avec raison que notre commission des lois a supprimé cette contrainte, qui s'apparentait à une immixtion dans la gouvernance des collectivités et à une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Il semble que l'Assemblée nationale ait oublié cette équation. Comme l'ont souligné les rapporteurs, le rôle du législateur n'est pas de faire peser une charge attentatoire à la libre administration des collectivités, qui relève de surcroît du domaine réglementaire. Plutôt que de contraindre, il convient de sensibiliser les collectivités territoriales et de faire confiance à l'intelligence territoriale. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'y a rien à ajouter

Le lien entre prévention de la délinquance et sécurité est au centre des attentes des Français à l'égard de l'État, mais aussi de leurs élus locaux.

Force est de constater que le bilan de ce dispositif est très positif. C'est pourquoi nous souhaitons que toutes les communes intègrent un conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, bien même elles n'ont pas l'obligation, qui a été abaissée de 10 000 à 5 000 habitants par cet article, de se doter d'un tel conseil à l'échelle de la commune. Ces conseils locaux remplissent des fonctions essentielles, notamment en matière d'information entre les forces de l'ordre, les acteurs sociaux, les acteurs de prévention de la délinquance, qui n'ont pas forcément spontanément le même regard sur les problèmes de sécurité. Si les séances plénières peuvent apparaître à certains acteurs comme un exercice de présentation et de communication, les groupes de travail et d'échange d'informations, en principe temporaires et thématiques, sur les violences faites aux femmes, sur la sécurité routière, sur les addictions, ont démontré leur utilité. Leur succès s'explique principalement par le fait qu'ils permettent cet échange. Le caractère vertueux de ces conseils locaux justifie que leur déploiement s'inscrive dans une logique de basculement d'un monopole central de l'État en matière de sécurité à une coproduction de sécurité à l'échelle locale entre les préfets et les élus locaux.

tout aussi soucieux que la plupart d'entre nous de la libre administration des collectivités territoriales. Nous proposons néanmoins de réinstaurer l'affectation

Instance clé de la prévention, le CLSPD exerce le pilotage de la politique locale de prévention de la délinquance. Il définit des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. Son efficacité doit être saluée dans la mobilisation de partenariats entre les différents acteurs de la société civile et des instances locales pour prévenir le basculement des jeunes dans la délinquance. C'est bien dans ce rôle que certains conseils, par manque de moyens humains, rencontrent des difficultés de coordination entre les différents acteurs de la commune et perdent de ce fait en efficacité. Le rapport d'information sur la refondation des CLSPD des députés Peu et Rebeyrotte pointe le nombre insuffisant des coordonnateurs. Ainsi, sur les 805 CLSPD qui existaient en 2018, seuls 574 coordonnateurs étaient recensés. Nous pensons que que l'affectation d'un agent public territorial au suivi, à l'animation et à la coordination des travaux du CLSPD ne pourra que renforcer l'efficacité de ce conseil si utile pour nos territoires.

pour renforcer le dispositif, tant la question du lien entre sécurité publique et prévention de la délinquance devrait être au coeur des politiques de sécurité publique. Cette proposition de loi prévoit beaucoup d'autres contraintes qui soulèvent beaucoup de problèmes.

majeurs, qui, hélas, se retrouvent parfois dans des comportements délictueux. Ces amendements sont donc centraux, car, si nous plaidons pour la répression des actes délictueux, la prévention doit être la règle, et elle devient de plus en plus urgente, vu la montée de la violence chez les très jeunes. Très bien

Lors de l'examen du texte en commission des lois, le rapporteur a supprimé l'article 30, qui donnait une base légale aux groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD). Un rapport parlementaire sur l'évolution et la fondation des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance des députés Peu et Rebeyrotte souligne l'utilité de ces GLTD dans le développement d'une justice de proximité de proximité que nous appelons de nos voeux. Ces structures d'échanges ont toute leur utilité pour renforcer la prévention et la lutte contre la délinquance dans les quartiers défavorisés. Par conséquent, le présent amendement du groupe Écologiste- Solidarité et Territoires vise à réintroduire l'article 30.

constitue, avec les dégradations et les incivilités, l'une des causes majeures des problèmes de troubles de voisinage et d'atteinte à la jouissance paisible que subissent les locataires. Les bailleurs sont souvent démunis face à ces situations, le problème étant le plus souvent d'apporter la preuve de ces trafics et des troubles que cela occasionne. Ces situations créent très souvent un climat de peur chez les locataires, qui n'osent témoigner par crainte de représailles. En parallèle, ces mêmes locataires ne comprennent pas l'inaction du bailleur, qui, en raison de l'insuffisance de preuves, ne peut engager d'action au fond en résiliation de bail. Le fait de pouvoir arguer de la condamnation pénale passée en force de chose jugée pour trafic de stupéfiants du locataire ou de l'un des occupants de l'un des occupants du logement hébergé comme motif automatique de résiliation du contrat de location permettra aux bailleurs d'engager plus facilement des actions contentieuses pour le bien commun des locataires souffrant de ces situations d'une particulière gravité et, ainsi, respecter leur obligation de faire cesser les troubles prévus à l'article 6-1 de loi du 6 juillet 1989.

Ce rapport examinerait l'opportunité de réinstaurer le code de déontologie de la police nationale entré en vigueur en 1986. S'agissant d'une demande de rapport, je crains que cet amendement ne soit rejeté ... Quel est

Le fait de vouloir changer l'intitulé de la loi après toutes les critiques venues de la société, c'est un peu la signature du crime, si je puis m'exprimer ainsi à propos de sécurité

des forces de sécurité intérieure présentes partout sur le territoire, dans toutes leurs missions régaliennes : la police judiciaire, le maintien de l'ordre, le renseignement et la sécurité publique, avec des missions claires et des moyens garantis. J'ai d'ailleurs relevé des élans droitiers très autoritaires et sécuritaires : il ne faudrait pas oublier que 12 000 à 15 000 postes de policiers ont

les forces de sécurité privée, avec le dévoiement de leurs missions de médiation, de proximité, de tranquillité, pour faire ce que l'État ne sait pas, ne peut pas ou ne veut plus faire. Nous finissons avec un texte en peau de léopard : des inégalités territoriales, puisque tout le monde ne pourra pas faire partout la même chose, et une forme d'illisibilité pour les citoyens dans l'accès au service public de la sécurité. Un autre aspect nous pose problème sur le fond. On observe un virage vers un nouveau paradigme qui met en danger certaines libertés,

Par diverses mesures, ce texte vise à donner des gages aux forces de l'ordre. Une fois encore, nous regrettons profondément que les pouvoirs publics s'engagent sur une voie toujours plus répressive et optent pour des moyens accrus de surveillance sans concertation avec la société civile ni égard pour le respect des droits fondamentaux, d'autant que de telles mesures ne participent pas directement à la lutte contre le terrorisme. Nous avons essayé de faire en sorte que

d'éviter les bavures policières. Je crois que nous n'y sommes pas du tout parvenus. Nous le déplorons également. Le point positif du texte a été la création, quasiment historique, d'une police municipale à Paris. En cette période de pandémie, où des dizaines de milliers de personnes sont contaminées, où des milliers sont décédées et où l'on craint le pire, un tel texte ne fait que rendre le climat plus anxiogène encore.

Dans un pays qui a mal géré la crise sanitaire, qui manque de vaccins et où la précarité ne fait que croître, avions-nous besoin de consacrer tant de temps

Selon nous, cette société présente le plus grand des dangers : celui d'un étouffement de nos libertés publiques, toujours plus asphyxiées par les lois sécuritaires qui s'accumulent sans cesse. Ces libertés- faut-il le rappeler ici ? -, nous les avons acquises à travers les siècles, au prix de luttes parfois difficiles.

projet de société est néfaste, nuisible. Il évoque les pires prédictions, jusque-là restées au rang de fictions ! Notre société doit rester ce qu'elle prétend être : une démocratie libre ! Et les dérives policières, dont la source réside dans une chaîne de commandement défaillante, doivent être combattues Nos amendements sur la police de proximité ou les contrôles au faciès ont été jugés irrecevables au titre de l'article 45. Disons plutôt qu'ils ont tout

Les autres dispositions du texte me semblent tout à fait pertinentes. Celles qui concernent l'encadrement de la sécurité privée contribueront à assainir le secteur. Celles qui déterminent le cadre de la vidéoprotection sont nécessaires ; elles permettront aux forces de l'ordre d'utiliser de nouvelles technologies tout en respectant la liberté publique. Enfin, il faut renforcer la protection de ceux qui nous protègent. Nos forces de l'ordre ne doivent pas être la proie des réseaux sociaux ni d'attaques délibérées. Notre groupe votera ce texte. La parole est à M. Philippe Mouiller,

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement sollicite du Sénat l'inscription à l'ordre du jour du jeudi 25 mars 2021, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention. Nous pourrions inscrire ce texte à l'issue de l'examen en deuxième lecture de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, et fixer la durée de la discussion générale à quarante-cinq minutes. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé.